4 % et 8 % des émissions nationales. Ces émissions sont en quasi totalité importées : la production des principes actifs des médicaments consommés en France est presque exclusivement localisée en Inde et en Chine, où les normes environnementales sont extrêmement souples. Le rapport de la mission sur la régulation des produits de santé remis à la Première ministre fin août l’annonçait : la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la consommation française de produits de santé ne pourra passer que par une intégration des enjeux environnementaux

? Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureuse d’être en votre compagnie ce matin.

rapporteure : défavorable. La prise en compte de l’empreinte carbone poserait un problème d’application pratique. Les industriels ne sont actuellement pas en mesure de fournir des données comparables et vérifiables, faute de méthodologie et de références partagées pour calculer leur empreinte. Je mets aux voix

: La parole est à Mme Anne Souyris. Le Comité économique des produits de santé (CEPS) est principalement chargé par la loi de fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel, ainsi que des prestations prises en charge par l’assurance maladie obligatoire.

ce rapport est riche et ses informations fort utiles. Assurer sa publication au plus tôt est un objectif partagé par de nombreux acteurs. Cependant, les informations contenues dans ce rapport ne sont pas

est de sécuriser l’ouverture de la possibilité d’un fractionnement des paiements de certaines thérapies innovantes, au lieu d’un paiement unique concomitant au traitement. En effet, cette faculté pourrait rendre acceptables des prix très élevés et provoquer une inflation des coûts de traitement. Un gouvernement peu

concernant la négociation du prix et des remises appliquées aux médicaments les plus onéreux. Or certaines de ces informations sont protégées par le secret des affaires. Leur caractère confidentiel renforce d’ailleurs les capacités de négociation du CEPS. Quel est l’avis du

Faute de transparence, il est difficile de distinguer la part des investissements publics et privés dans le développement d’une nouvelle molécule. Cet amendement vise à assurer une réelle transparence sur les montants des investissements publics de recherche et de développement bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments.

de médecine au Collège de France. Selon lui, plusieurs publications montrent que les bénéfices du secteur pharmaceutique sont plus importants que ceux de tous les autres secteurs industriels. Dans les plus grandes entreprises mondiales, les dépenses de marketing dépassent largement les dépenses de recherche et de développement. concernant les dividendes distribués et les rachats d’actions. On parle de 7 % à 8 % de rentabilité. De plus, une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics. L’exemple du Zolgensma est explicite : mis au point avec la contribution du laboratoire de l’AFM

l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

pris en charge ou ayant vocation à l’être. Or l’obtention de ces montants nécessite une comptabilité analytique complexe à mettre en œuvre. En outre, cette donnée n’est pas toujours la plus

avec les coûts de production des laboratoires pharmaceutiques. À titre d’exemple, entre 2004 et 2017, le coût de prise en charge du mélanome métastatique a été multiplié par 165 en France.

exploitant certains médicaments doivent mettre à la disposition du CEPS le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié. Nous souhaitons désormais aller plus loin en imposant au CEPS de tenir compte des investissements publics lors de ses négociations avec les laboratoires pharmaceutiques sur la fixation des prix

soutenabilité économique des médicaments anticancéreux onéreux, l’Académie nationale de médecine appelle ainsi à mettre en place une production publique de traitements anticancéreux personnalisés. Ainsi, à Barcelone, une production publique de cellules a permis de réduire le coût d’une thérapie à 89 290 euros contre 320 000 euros dans le privé. De la même manière, concernant les anticancéreux protégés par brevet, l’Académie préconise dans son rapport de créer, comme aux États Unis, une structure à but non lucratif acquérant les traitements pour approvisionner les hôpitaux à prix fixe, quel que soit le volume.

et aux coûts de recherche, de développement et de commercialisation réellement supportés par les industriels. Cette opacité, qu’a dénoncée la commission d’enquête sénatoriale sur la pénurie de médicaments, est également constatée par l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament,

Aucun critère légal de fixation du prix du médicament ne tient compte des coûts de production de celui ci pour le laboratoire qui l’exploite. Cette situation présente l’avantage, si je puis m’exprimer ainsi, de permettre la fixation du prix du médicament sans dépendre d’informations fournies fournies par l’industriel, qui se révéleraient difficilement vérifiables ; mais elle présente l’inconvénient de permettre la rémunération, financée par l’assurance maladie, d’une innovation thérapeutique à un prix dépassant largement le coût de production.

pour les industriels. En 2019, le législateur a tenté de renforcer la transparence en la matière en contraignant les entreprises à rendre public le montant des investissements publics de recherche et de développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits sur la liste en sus Ces dispositions n’ont toutefois pas eu l’effet escompté, en raison du périmètre restreint des informations attendues, mais aussi parce que le CEPS n’est pas en mesure de les contrôler. C’est pourquoi nous proposons de renforcer la transparence dans le domaine du médicament en rendant obligatoire, au delà d’un certain niveau de prix revendiqué,

et de prise en charge financière par l’assurance maladie. C’est le cas du Paxlovid et du Beyfortus. Pourtant, aucune information n’est publiée sur les prix de ces médicaments achetés en centrale,

sur l’amendement n° 779 rectifié – lui permettant chaque année d’instruire les données et les dispositions votées dans les PLFSS successifs. En revanche, la transmission chaque année de données concernant les commandes de l’État et de Santé publique France,

observe une forte progression des dépenses des hôpitaux pour les médicaments inscrits sur la liste en sus. En 2021, cette dépense représente 5,7 % de la consommation hospitalière et se concentre sur un faible nombre de médicaments et de dispositifs médicaux.

En effet, la multiplication des dispositifs médicaux numériques appelle à en différencier les apports pour les patients et à revaloriser ceux qui font plus largement évoluer le confort de vie lors d’une affection de longue durée (ALD), qui, par définition, a un impact durable sur la vie quotidienne du patient.

Ainsi, par cet amendement, nous entendons revaloriser cet impact sur la vie quotidienne des patients, en l’appliquant aux remboursements de ces produits. Puisque cette proposition ne vise qu’à faire évoluer la pondération des critères de modulation de la base forfaitaire, elle n’entraîne pas de charge supplémentaire pour la sécurité sociale.

Il s’agit d’ouvrir aux dispositifs médicaux inscrits en ligne générique, et non seulement à ceux qui sont inscrits sous nom de marque, la disposition permettant la prise en compte dans la tarification de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation nationale des sites de production. la commission sur l’amendement

chers collègues, j’aimerais appeler votre attention sur une maladie particulièrement présente en outre mer, la dengue. La dengue peut provoquer chez les personnes qui la contractent des complications graves, voire fatales. Les conséquences sont à la fois physiques et mentales – ces dernières pouvant Une épidémie de dengue, c’est un engorgement des centres de santé difficile à juguler et des touristes forcément moins nombreux, avec les répercussions socioéconomiques que l’on peut imaginer. Nous observons chaque année une augmentation du nombre de cas ; les perspectives ne sont d’ailleurs pas bonnes,

du régime temporaire de prise en charge de certains médicaments en fin d’accès précoce. Il convient de prévoir une implication directe et immédiate de ce régime sans attendre la publication d’un décret d’application et d’éviter ainsi les ruptures de prise en charge et les pertes de chances qui en découlent pour les personnes malades concernées. Cet amendement vise également à fixer un cadre contractuel permettant de préciser l’engagement des industriels à approvisionner le marché afin de sécuriser l’accès des patients au traitement et d’éviter qu’ils puissent être pris en otage par ces mêmes dans l’hypothèse où l’évaluation de leurs produits par la Commission de la transparence ne satisferait pas leurs attentes ou leurs exigences. Quel commission ? L’amendement n° 927 vise à ajouter un caractère contractuel à l’engagement d’approvisionnement approprié et continu pour les spécialités en accès précoce. Sur le principe, la commission est bien sûr favorable à ce que les industriels du médicament assurent, en contrepartie du bénéfice de l’accès précoce, un approvisionnement suffisant du territoire national, et ce dans l’intérêt des patients. Toutefois, ce point étant véritablement technique, la commission sollicite l’avis du Gouvernement. l’avis du Gouvernement.

telle mention ne semble ni nécessaire ni opportune, dans la mesure où les obligations d’approvisionnement ont un caractère légal et réglementaire. De plus, le terme « contractuel » pourrait laisser penser qu’il est possible

l’amendement n° 297 rectifié. Au regard des enjeux d’accès aux traitements et de maintien de l’innovation en France, cet amendement vise à simplifier les modalités de fixation de l’indemnité à laquelle la spécialité sera prise en charge par l’assurance maladie lors de la période de prise en charge temporaire. à supprimer la mention de prix européen le plus bas initialement prévue et à maintenir comme seule référence l’indemnité libre demandée par le laboratoire pour cette spécialité, à laquelle sera appliqué un mécanisme de décote défini par voie réglementaire. Cette décote ne concernera toutefois pas les médicaments disposant, sur une autre indication, d’un prix ou d’un tarif fixé au titre de la liste en sus et de la liste en officine, ni ceux auxquels s’applique, sur une autre indication, un prix maximal de vente aux établissements de santé. travers de cet amendement, c’est une solution équilibrée pour la fixation des paramètres de calcul du niveau de l’indemnité de prise en charge temporaire qui est retenue. En effet, s’il est certain que cette indemnité doit prendre en compte les résultats insuffisants obtenus par la spécialité lors de sa première évaluation et ne saurait donc être maintenue au niveau qui prévalait lors de la période d’accès précoce, il n’en est pas moins évident qu’une prise en charge insuffisante priverait le dispositif de toute attractivité, ce qui nuirait, en dernier ressort, aux patients.

à Mme Émilienne Poumirol. Cet amendement vise à préciser que l’entreprise pharmaceutique qui va cesser la production d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), en particulier un générique, est mise en demeure de trouver un repreneur.

dans la mesure où l’information de l’ANSM produit un effet juridique concret, à savoir le début du délai de neuf mois imparti pour la recherche d’un repreneur et les justifications liées. J’ai cependant considéré que la suite de la rédaction de l’article ne souffrait pas d’ambiguïté

est à Mme la rapporteure. En cas d’absence de reprise de la commercialisation par une autre entreprise, l’exploitation et la fabrication pourraient être confiées à un établissement pharmaceutique public. Cependant, la reprise de cette production pourrait n’être organisée qu’à l’issue d’un délai de neuf mois, soit moins de trois mois avant l’arrêt possible de la production par l’entreprise par l’entreprise qui l’exploite. Par conséquent, il convient de prévoir l’information des établissements pharmaceutiques susceptibles d’assurer la reprise de l’exploitation ou de la fabrication, en vue de leur permettre d’anticiper l’organisation de celle ci avec les façonniers.

le titulaire de l’AMM doit également informer les établissements pharmaceutiques détenus par une personne morale de droit public. Ce faisant, il s’agit de faciliter l’éventuel transfert de l’exploitation ou de la fabrication du médicament à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public satisfaisantes. Reste que ces établissements n’ont vocation qu’à reprendre en ultime recours certains produits définis au cas par cas par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

mois à six mois. En effet, nous considérons que, compte tenu de l’augmentation croissante du nombre de pénuries de médicaments et de la nécessité d’assurer la continuité de la production des médicaments concernés, nous ne pouvons laisser des délais trop importants pour fournir un tel rapport. La politique du médicament ne peut

Un délai de six mois ne paraît ni raisonnable ni cohérent avec le souci de démarches qualitatives et avec les échanges nécessaires entre l’exploitant et les repreneurs potentiels. Ce délai raccourci pourrait même être contre productif, limitant l’effort de recherche qui, au bout de six mois, ne serait plus contrôlé. Si nous voulons que ce dispositif ait un sens, il faut que les conditions d’application soient raisonnables et cohérentes avec les réalités des entreprises. En outre, le raccourcissement du délai accélérerait de fait la reprise par l’établissement public six mois avant l’arrêt théorique de la production. Ce transfert pourrait donc intervenir dans un délai insuffisant pour permettre à l’établissement

d’imposer des contraintes aux laboratoires pharmaceutiques sont rejetés. Or nous ne sommes pas là pour défendre l’industrie pharmaceutique ! Nous sommes là pour défendre notre population,

Nous devons avoir comme préoccupation la santé publique et l’intérêt de nos concitoyens.

depuis 2018. Obliger les entreprises à trouver un repreneur est un premier pas que nous saluons, mais ce n’est pas suffisant. Nous devons contraindre davantage les entreprises pharmaceutiques et les sanctionner lorsqu’aucun repreneur n’a été trouvé. L’accès de la population aux médicaments

leur qualité de vie, voire, parfois, leur survie. C’est pourquoi nous proposons une sanction à l’égard des entreprises qui n’ont pas trouvé de repreneur, à hauteur de 3 % de leur chiffre d’affaires annuel. En sanctionnant les entreprises pharmaceutiques qui retirent un médicament sans avoir trouvé

que les entreprises « assurent un approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France ». Il est difficile d’imaginer que les entreprises se satisfassent des ruptures d’approvisionnement. Cette nouvelle obligation de garantir

Les études ou essais cliniques susceptibles d’être défavorables au développement commercial ou au remboursement des spécialités pharmaceutiques ne sont pas publiés, voire sont interrompus ou pas même engagés.

autorise des demandes sans fondement scientifique. L’amendement tend par ailleurs à prévoir que l’inscription sur la liste des médicaments remboursables est conditionnée à une évaluation du médicament et au suivi de son efficacité.

aux thérapies accessibles, certaines formes d’épilepsie sévères et pharmacorésistantes, certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou à ses traitements, des situations palliatives et la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou d’autres pathologies du système nerveux central. La

l’expérimentation du cannabis médical prévue par la loi de financement de la sécurité sociale de 2019. Cet amendement vise à préciser la marge de manœuvre du Gouvernement dans la détermination de la liste des maladies pour lesquelles le cannabis pourrait dorénavant être prescrit. Il tend à prévoir que l’arrêté qui fixera la liste des indications thérapeutiques se borne à reprendre lors de l’expérimentation de 2019, à savoir les cinq indications suivantes : douleurs neuropathiques réfractaires aux traitements existants, certaines formes d’épilepsie, certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou à ses traitements, les soins palliatifs et la spasticité spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou d’autres pathologies du système nerveux central. Néanmoins, nous soutenons la généralisation du cannabis médical pour d’autres applications amorcée dès à présent

Par cet amendement, supprimons l’obligation de mise en place par le détenteur de l’autorisation du recueil des données de suivi des patients traités et garantissons le respect de la vie privée, du secret médical et des données de santé. Quel est l’avis de la commission ? Il est ? Il est défavorable, madame la présidente. Le suivi un recueil de données des patients traités, à la charge de l’exploitant, contribuera à la surveillance des médicaments à base de cannabis qui ne bénéficieront pas, dans le dispositif proposé, d’une autorisation de mise sur le marché.

notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui encadrent la collecte et la conservation des données à caractère personnel et exigent le consentement préalable de la personne concernée. La mise en place de dispositifs de suivi sécurise le développement de nouveaux médicaments et, surtout, ne limite pas l’exercice

L’utilisation du cannabis thérapeutique doit être accompagnée d’une formation des professionnels de santé. Cette formation doit rester encadrée par le cadre législatif du régime général des médicaments et et ne doit pas faire l’objet d’une politique d’information plus stricte, afin de convaincre les professionnels de se former à cette question et d’intégrer le programme national de cannabis à visée médicale. Le cannabis thérapeutique doit relever du régime général. Cet amendement vise à supprimer les restrictions quant à l’information des professionnels de santé. Les rapports successifs réalisés par le Gouvernement, le rapport d’étape présenté par le Parlement en octobre 2022 et les documents fournis en 2023 montrent l’importance de la mobilisation des professionnels de santé dans l’expérimentation du cannabis thérapeutique. Les enjeux sont doubles un plus grand nombre de professionnels de se former sur le cannabis thérapeutique, mais aussi de contrôler et de limiter l’influence des entreprises du cannabis thérapeutique sur les professionnels. Il est donc souhaitable que cette responsabilité revienne à l’ANSM, qui décidera de la marge de manœuvre des sociétés privées. Quel

cours. L’article 36 prévoit déjà la possibilité pour le Gouvernement de saisir la HAS en vue d’une éventuelle prise en charge de ces médicaments par la collectivité. Une telle saisine sera articulée avec le travail d’expertise en cours à l’échelon européen.

En l’état actuel du droit, cette continuité n’est pas garantie, puisque le bénéfice de l’assurance maladie est conditionné à la résidence « stable et régulière » en France. D’une part, cette condition a pour conséquence que les personnes qui déménagent à l’étranger perdent, sauf cas particulier, leur couverture par l’assurance maladie ; d’autre part, la condition d’un séjour « stable et régulier » a pour conséquence qu’une personne qui revient en France après avoir vécu à l’étranger

l’étranger. Ce délai de carence les expose à des risques sanitaires et financiers importants. Pour y remédier, il convient de garantir immédiatement à toute personne qui revient de l’étranger le bénéfice d’une prise en charge de ses frais de santé.

de bénéficier de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité dès leur retour en France. Entrée en vigueur le 1 janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMa) permet à toute personne travaillant en France ou, si elle n’exerce pas d’activité professionnelle, à toute personne résidant en France de manière stable et régulière d’être affiliée au régime français. Pour justifier de la stabilité de sa résidence en France, une personne n’exerçant pas d’activité professionnelle et souhaitant s’affilier à l’assurance maladie française doit produire un justificatif démontrant qu’elle réside bien en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Certaines catégories de personnes listées à l’article D. 160 2 du code de la sécurité sociale n’ont pas à justifier de cette condition. Aussi, bien que les anciens assurés du régime français ne soient pas mentionnés en tant que tels dans cet article du code de la sécurité sociale, plusieurs solutions peuvent leur être apportées en fonction de leur situation. Soit, comme vous le mentionnez, l’assuré exerce une activité professionnelle à son retour en France

ininterrompue depuis plus de trois mois en France ; dans ce cas, le membre de la famille qui l’accompagne ou le rejoint peut s’affilier immédiatement auprès de la caisse primaire d’assurance

pendant les trois premiers mois de son séjour en France. C’est ce que prévoient d’ailleurs les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale. Cette personne peut alors utiliser la carte européenne d’assurance maladie en France pendant cette période et s’en prévaloir pour s’affilier à la PUMa. Soit la personne s’est affiliée, le temps de son expatriation, auprès de la Caisse des Français de l’étranger (CFE). Dans ce cas, la CFE prévoit également un maintien de droit lors du retour en France. Soit la personne ne conserve aucun droit de son précédent régime, ne travaille pas en France et n’y réside pas depuis au moins trois mois. Elle

d’un régime français puissent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé dès leur retour en France et sans délai de carence. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement

et autonomie. Nous sommes inquiets face à l’immensité des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous en connaissons les conséquences sur les établissements d’accueil des personnes âgées, notamment publics, et sur les collectivités territoriales, qui en sont les gestionnaires. Les soignants, comme les gestionnaires, n’en peuvent plus. En Bretagne, des élus se sont organisés pour nous alerter – vous alerter, madame la ministre en créant un collectif. Des crédits supplémentaires ont été inscrits pour tenter de colmater les déficits. Je ne sais s’ils suffiront, mais ce dont je suis sûre, c’est que ces crédits permettront seulement de répondre ponctuellement aux difficultés financières des établissements, qui ne peuvent plus payer leurs factures d’énergie ni leurs charges de personnel. Le problème est structurel : quel reste à charge pour les familles ? Quelle contribution pour les collectivités ? De nombreuses réflexions ont été menées

Cet amendement, rédigé avec ma collègue Monique Lubin, vise à supprimer l’article 37. En effet, cet article met en place une simplification du mode de financement des Ehpad et des en fusionnant à compter de 2025, dans les départements volontaires, les dépenses afférentes à la prise en charge de la dépendance et celles afférentes aux soins, en les regroupant dans une section unique relevant d’un financement par la cinquième branche de la sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité se distingue par son caractère irréversible pour les départements qui s’y engageraient. C’est un premier problème. Elle induit également, pour les départements, une modification de la gouvernance de la politique locale de la dépendance et de l’autonomie dans une direction qui pourrait rendre impossible toute action volontariste, innovante et d’ampleur en la matière de la part de ces collectivités, qui exercent aujourd’hui cette compétence. Cette modification met également en péril l’existant. C’est pourquoi le présent amendement tend à supprimer l’article

En effet, cette répartition perd de sa pertinence compte tenu de l’évolution du profil des résidents, qui sont de plus en plus dépendants. Par ailleurs, ce modèle de financement entraîne des coûts de gestion importants pour les établissements. Les variations du forfait dépendance d’un département à l’autre peuvent engendrer des inégalités territoriales. Enfin, le coût induit pour les départements est également élevé, au regard de leur marge de décision spécifique. La grande majorité des établissements soulignent la nécessité d’une réforme et considèrent que le fait d’avoir affaire à un financeur unique est une priorité. Or il semble plus cohérent que ce financeur soit la branche autonomie et que le pilote soit l’ARS. Le département conserverait néanmoins un rôle important à l’égard des Ehpad outre ses compétences d’autorisation des établissements et d’aide sociale à l’hébergement, il jouerait notamment un rôle de coordination. La commission est donc favorable à l’engagement d’une réforme structurelle en ce sens. En revanche, comme vous le soulignez, le dispositif proposé est problématique en ce qu’il institue une mesure pérenne à la carte. Je vous présenterai dans quelques instants

irréversible de la mesure. Aussi, nous pourrons transformer la fusion des sections en une expérimentation plus encadrée, afin de disposer d’une évaluation solide et de rassurer les départements qui sont prêts à franchir le pas.

pertinente pour les résidents et leur famille Cet amendement tend à réécrire l’article 37 pour mettre en place une expérimentation croisée, d’une part du pilotage de la section dépendance par les ARS, d’autre part du pilotage de la section soins par les départements.

symétrique pour les ARS et les départements. Sur la forme, contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs, les modifications législatives que vous proposez ne comportent pas de dispositions relatives à une fusion des sections tarifaires soins et dépendance, comme cela est envisagé. Le texte propose seulement une mesure de réciprocité pour la fixation du forfait soins, qui pourrait être confiée aux départements et pour la fixation du forfait dépendance, qui, inversement, pourrait être confiée aux ARS.

est à Mme le rapporteur. La fusion des sections soins et dépendance pour le financement des Ehpad comporterait de nombreux avantages pour les établissements et rendrait le système plus lisible pour l’ensemble des acteurs. Toutefois, la mesure proposée à l’article 37, qui est à la fois pérenne et facultative, pourrait paradoxalement créer des complexités supplémentaires et laisser s’installer dans la durée des disparités plus profondes entre les départements. Cet amendement vise donc à transformer cette mesure en une véritable expérimentation, qui pourrait être déployée sur une durée de trois ans, à compter du 1 janvier 2025, dans un maximum de dix départements volontaires. Cette expérimentation donnerait lieu à une évaluation par la CNSA et à la remise au Parlement, six mois avant son terme, d’un rapport envisageant les conditions de sa pérennisation et de sa généralisation.

les modalités de la réforme, mais à chaque département d’en mesurer les impacts pour lui même. À titre d’exemple, le vice président de la métropole de Lyon, que j’ai consulté, estime qu’il ne sera pas possible pour sa collectivité de s’engager dans le dispositif de fusion prévu si la date butoir du 31 mars 2024 est maintenue.

Les financements ne sont pas à la hauteur. Vous avez créé une cinquième branche, mais elle n’a pas de feuilles… Finalement, on en est réduit à gérer l’accueil des personnes âgées avec des bouts de ficelle

frais de séjour par leurs revenus courants. Le séjour en établissement est coûteux pour tous, mais il est totalement insoutenable pour les plus modestes. Le système actuel est d’ailleurs peu justifié : d’une manière générale, les plus modestes ne sont pas aidés à la hauteur de leurs besoins ; les ménages modestes sont moins aidés que les plus aisés.

que le reste à vivre des résidents des Ehpad dans les départements qui fusionneront leurs sections « soins » et « dépendance » sera défini après avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

à des séjours qui, au demeurant, ne sont la plupart du temps pas choisis, mais subis ». Or, parmi les résidents en Ehpad, les personnes âgées pauvres, fragiles et isolées sont nombreuses. Elles sont confrontées à des taux d’effort considérables : seulement une petite partie

mais il est parfaitement insoutenable pour les plus modestes. Le système actuel est par ailleurs peu justifié : globalement, les plus modestes ne sont pas aidés à la hauteur de leurs besoins ; les ménages modestes sont moins aidés que les plus aisés. aisés. » Selon ce même rapport, « il est donc possible, en établissement comme à domicile, de demander à chacun de contribuer selon ses moyens et d’être soutenu selon ses besoins ». Tel est l’objet de notre amendement.

Mes chers collègues,

précédents. Les amendements identiques n 1029 et 1193, qui prévoient une concertation avec le président du conseil départemental sur le montant du forfait unique pour les soins et la dépendance, semblent contraires au principe de l’expérimentation c’est bien un pilotage par l’ARS qu’il s’agit d’expérimenter, étant entendu que les départements conserveront, pour leur part, la compétence de l’aide sociale à l’hébergement. l’hébergement. L’amendement n° 1190 prévoit un avis de l’Assemblée des départements de France sur les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique il va de soi que, pour que le dispositif fonctionne, les départements doivent être associés à son élaboration. L’amendement n° à imposer la prise en compte des ressources des résidents dans la fixation de leur participation journalière, est satisfait : il sera garanti aux personnes accueillies un montant minimal laissé à leur disposition.

vise à ce que les ressources des résidents soient prises en compte pour fixer leur contribution à la future section unique « soins et entretien de l’autonomie ». Lors du passage au forfait unique, la participation des résidents deviendra forfaitaire et sera uniformisée,

Par ailleurs, la mise en œuvre d’une gestion en fonction des ressources est d’une grande complexité, on le sait, pour les Ehpad. Ce mécanisme irait donc à rebours de la simplification qui est justement recherchée.

il s’avère qu’une telle mesure devrait nécessairement s’accompagner du transfert d’autres compétences actuellement détenues exclusivement ou conjointement par les ARS

l’expertise en matière de circuit du médicament ; la coordination entre le sanitaire et le médico social, etc. En résumé, cette mesure soulève ainsi de nombreuses interrogations très concrètes dans de nombreux des domaines : est ce que les départements discuteront désormais de l’organisation d’une pharmacie à usage

vendredi dernier, l’assemblée générale de la Fédération hospitalière de France pour la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur. J’ai été étonné de constater que tous les médecins coordonnateurs et tous les directeurs d’Ehpad souhaitent l’instauration d’un financeur unique. Et tous,

Les prestations historiques de l’hébergement pourront alors être recentrées sur le gîte et le couvert. Les prestations à visée socio éducatives et ludiques, quant à elles, pourraient ainsi être reversées dans la section « soins et dépendance

l’avis de la commission ? Vous entendez priver de financement public les établissements dans lesquels la rémunération de certains salariés ou associés dépasse neuf fois la rémunération moyenne au sein de l’établissement. Certes, améliorer le partage de la valeur dans le secteur du grand âge serait bénéfique pour la reconnaissance de ces personnels et l’attractivité de ces métiers. Toutefois, la commission a estimé que le plafonnement de la rémunération des dirigeants n’était pas la bonne méthode pour le garantir. L’avis est défavorable.

La compensation des revalorisations du Ségur a par exemple été calculée en prenant en compte les dispositifs d’allégement de charges, différents d’un secteur à un autre. De façon générale, la tarification des établissements et services médico sociaux tient compte des mesures catégorielles de la fonction publique ou des évolutions salariales parfois différentes liées aux conventions collectives pour le secteur privé à but non lucratif. Je suis défavorable à ces trois amendements

également des pistes pour rétablir les conditions d’un versement effectif de la rémunération des personnels concernés et pour assurer, plus largement et durablement, l’attractivité de tous ces métiers. En effet, en 2022, certaines professions du soin et des secteurs social et médico social étaient éligibles éligibles aux mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé et des accords Laforcade. Or nombre d’établissements et services sociaux et médico sociaux ont annoncé n’avoir pas reçu de leur autorité de tarification et de contrôle les crédits correspondants.

En 2022, certains professionnels des domaines sanitaire, social et médico social étaient éligibles aux mesures de revalorisation du Ségur de la santé et des accords Laforcade. Cependant, de nombreux établissements et et services sociaux et médico sociaux ont signalé ne pas avoir reçu les crédits correspondants de leurs autorités de tarification et de contrôle. Les professionnels de ces établissements participent pourtant pleinement à une mission d’intérêt général essentielle dans un contexte de vieillissement de la population.

également des recommandations pour établir une revalorisation effective des rémunérations du personnel concerné, ainsi que pour améliorer durablement l’attractivité des métiers dans les secteurs sanitaire, social et médico social.

Confrontés à l’inflation et à l’augmentation de leurs charges, de plus en plus d’Ehpad publics se retrouvent en situation déficitaire : ils étaient 42 % en 2019, 80 % en 2022. Les circonstances sont donc plus critiques que jamais. Au delà de l’enjeu financier, nous faisons face à un défi de société. Nos aînés méritent de vivre dans la dignité. Les Ehpad publics jouent un rôle central à cet égard, en offrant des soins de qualité qui demeurent les plus accessibles possible. Préserver ce système serait le témoignage du juste respect que nous devons à nos aînés. Le rôle de l’État est justement d’assurer des conditions de vie décentes au plus grand nombre d’entre eux. Or, sans financement supplémentaire, les Ehpad publics ne pourront plus garantir le service et la qualité de soins qu’ils offrent actuellement. Nous risquons un effondrement du système. Par cet amendement, nous demandons donc la remise d’un rapport sur le financement des Ehpad publics, rapport nécessaire pour éclairer sur la situation en cours et proposer des solutions viables. Des recommandations concrètes pour améliorer ce financement

vis à vis des professionnels de la santé et du secteur médico social puissent être honorés. Un travail d’analyse des états réalisés des recettes et des dépenses pour 2022 des établissements et services médico sociaux, mené cet été en lien avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, permettra

au sein d’établissements et de services sociaux et médico sociaux, ainsi que de les transposer à la branche de l’aide à domicile (BAD) du secteur privé non lucratif. Pour cette dernière, l’avenant 43,

que soit remis un rapport sur le coût d’une extension du Ségur au personnel des services d’aide et d’accompagnement à domicile du secteur privé non lucratif, ainsi que sur une uniformisation des dispositifs de compensation.

L’activité d’aide et de soins à domicile se développe, du fait du vieillissement de la population, de la politique de réduction des séjours hospitaliers et, bien sûr, du virage domiciliaire. J’ai mené une petite enquête, qui m’a appris que certaines villes accordaient des forfaits de stationnement aux infirmiers, mais pas aux aides soignantes

Par ailleurs, les services de répit de longue durée pourraient être coordonnés avec les plateformes de répit autorisées par les ARS, dans l’objectif de réguler les demandes, d’offrir les prestations au public concerné et de contrôler la qualité des interventions et l’information

présentant un handicap ou une suspicion de handicap. Pour mettre en œuvre ce service, il conviendra de s’appuyer sur les mesures de repérage déployées par les acteurs

Pour garantir l’efficience du dispositif, il faut, d’une part, s’assurer que les moyens financiers et humains qui lui seront consacrés seront suffisants, en prévoyant notamment des effectifs suffisants de personnel qualifié, et, d’autre part, améliorer l’attractivité des métiers concernés par le dispositif.

faute d’un environnement scolaire inclusif, l’école demande encore trop souvent aux enfants en situation de handicap de s’adapter, au risque de les stigmatiser et,, de les exclure. Ce rapport souligne également le décalage entre, d’une part, la faible augmentation des moyens humains et financiers

du service de repérage, de diagnostic et d’accompagnement précoce. Il s’agit d’une avancée majeure pour les enfants présentant un handicap et, en particulier, un trouble du neuro développement (TND). Je souhaiterais toutefois relayer quelques interrogations qui méritent qu’on leur prête attention et que des précisions

pour les familles les plus démunies, comme c’est le cas actuellement dans les PCO. Enfin, il est urgent d’avancer sur les enjeux relatifs aux conditions de scolarisation de ces enfants, ainsi que d’améliorer le dépistage des troubles du neuro développement, l’accompagnement des personnes qui en sont atteintes, enfants comme adultes, et le répit de leurs proches aidants. La parole